amendement vise à étendre les mesures prévues par l'article 40 s'agissant de l'encadrement de la publicité en faveur des produits de santé au sein des établissements de santé à l'ensemble de ces établissements, y compris ceux qui relèvent du secteur privé ou du secteur privé non lucratif.

il y a une vingtaine d'années pour soigner les malades atteints du VIH. Elle permet, pour des raisons de santé publique, de contourner un brevet existant et de créer un médicament de même intérêt thérapeutique à un tarif abordable.

pas ? Le Gouvernement nous a invités, depuis le début de l'examen du PLFSS, à faire preuve d'innovation et à voter des pratiques

a établi que « le risque en cas de recours à la licence d'office est donc que le juge national impose à l'État de payer le prix demandé par le laboratoire, lequel prix viendra, du point de vue des finances publiques, s'ajouter au coût d'achat

la négociation conventionnelle et, jusqu'à présent, nous avons toujours réussi à aboutir à un prix négocié, acceptable pour la communauté. Mais peut-être aurons-nous un jour à nous servir de ce dispositif si nous n'aboutissons pas à un accord.

plus générale, de l'économie du médicament, de la phase de recherche à celle de commercialisation. On sait que l'opacité qui peut régner parfois nourrit des suspicions. C'est pourquoi nous proposons que soit rendu public le chiffre d'affaires par produit réalisé chaque année par les entreprises. L'accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel à la suite des diverses remises- taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance permettrait une vision éclairée, pour les parlementaires et la société civile, des finances publiques et de la politique publique du médicament. Actuellement, seul le montant global des remises est publié chaque année. Nous souhaitons aller plus loin dans cette transparence et améliorer la clarté concernant les dépenses de santé, afin de permettre une approche mieux informée de l'économie générale du médicament, de sa recherche à sa commercialisation. commercialisation. Cette transparence accrue est d'autant plus pertinente que le chiffre d'affaires réalisé peut, lorsqu'il dépasse un certain seuil, conduire au versement de contributions à l'assurance maladie par l'entreprise exploitant le médicament, ce qui entre en jeu lors de la fixation du prix de certains médicaments. On nous oppose régulièrement le secret des affaires.

Je pense réellement que l'adoption de votre amendement aboutirait à des négociations moins faciles pour le CEPS. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.

Derrière ce refus se cache, en fait, une forme d'anticipation de la fermeture des pharmacies minières, qui a permis d'accélérer l'ouverture de nouvelles officines libérales. Notre propos, je le dis très clairement, n'est pas d'opposer les unes aux autres. Ce qui est en jeu, c'est le traitement équitable des pharmacies minières. On en est loin : tout est fait, en effet, pour justifier et accélérer la fermeture des pharmacies du régime minier. la méthode comptable sépare les résultats très excédentaires de la vente du matériel médical des résultats globaux de l'officine minière, ce qui fragilise ces derniers. Madame la ministre,

qui ont été autorisées à recevoir les patients de tous les autres régimes. En fait, ces nouveaux patients n'ont contribué qu'à hauteur de 10 % à peu près du chiffre d'affaires des trois pharmacies,

L'article 41 met en place plusieurs mesures de régulation économique du secteur des dispositifs médicaux. Si leur philosophie peut aisément être partagée compte tenu du dynamisme des dépenses associées à ces dispositifs, il est à craindre que leur caractère ambitieux et soudain n'aboutisse à une déstabilisation profonde de ce secteur. Celui-ci est, en effet, en cours de structuration et repose encore principalement sur un réseau de petites entreprises produisant le plus souvent en petites séries et avec un gain marginal faible. En outre, la croissance des dépenses en matière de dispositifs médicaux et de prestations associées s'explique en partie par le développement des prises en charge ambulatoires, qu'il s'agit, par ailleurs, d'encourager. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif, en conservant les autres mécanismes d'ajustement prévus par l'article 41. Il sera toujours possible aux parties prenantes de convenir d'une mesure de régulation équivalente par voie conventionnelle.

de petite taille ou n'ont pas les capacités financières susceptibles de leur permettre d'absorber ces difficultés. Par conséquent, je souhaite à tout le moins que l'on mette à l'étude les conséquences

L'idée n'est absolument pas d'empêcher le virage ambulatoire. Il s'agit, dans l'hypothèse où l'utilisation d'un dispositif par un prestataire

que l'ambulatoire fait faire des économies. Sur le plan social, je voudrais juste m'attarder sur une catégorie de personnes chez qui l'hospitalisation peut être particulièrement délétère : je veux parler des personnes âgées.

le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionné aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7, des produits et prestations concernés. Ce nouvel outil de régulation sur les produits et prestations relevant de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie s'inspire des mécanismes utilisés pour le médicament. Il est, à notre sens, incompatible avec les spécificités du secteur de la santé à domicile. En effet, l'évolution démographique et épidémiologique conjuguée à une volonté politique forte en faveur du virage ambulatoire- ces sujets ont déjà été évoqués -conduit à une augmentation inéluctable du nombre de patients souffrant de maladies chroniques. L'objet de l'amendement est de garantir que, dans l'hypothèse où le CEPS fixe un montant maximal des dépenses de l'assurance maladie au-delà duquel une baisse de prix pourra être décidée, ce montant maximal ne soit pas uniquement au regard des critères posés par l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, mais prenne également en compte les facteurs de cette évolution, en lien avec la démographie, l'épidémiologie et la volonté politique d'un accroissement des prises en charge à domicile,

permettent ainsi aux syndicats de représenter l'ensemble des pharmaciens d'officine au sein des différentes autorités compétentes. Il semble donc inopportun, voire inutile, de permettre à quelques pharmaciens non représentatifs de venir défendre devant le CEPS leurs propres intérêts économiques. L'amendement

L'article 42 ajoute un nouveau cas de recours à la procédure de demande d'accord préalable, lorsque « le recours à une autre prestation est moins coûteux », ce qui est d'ailleurs quelque peu contradictoire avec les objectifs annoncés dans

de la sécurité sociale uniformise et renforce le mécanisme d'autorisation préalable du service de contrôle médical des caisses d'assurance maladie. Ce mécanisme conditionne la prise en charge, par l'assurance maladie, d'une prestation ou d'une prescription de produits par les praticiens. Cette extension de l'autorisation préalable s'inscrit pleinement dans les objectifs de réduction des dépenses de l'assurance maladie annoncés par le Gouvernement, car c'est bien le montant du coût qui conditionnera la prise en charge, ou non, d'une prestation ou d'une prescription. Dans le cas des médicaments, l'accord préalable de prise en charge par l'assurance maladie se base sur le prix unitaire du produit. Or il est de notoriété publique que certains médicaments, plus coûteux que d'autres- notamment les nouvelles molécules -, offrent de meilleurs résultats, épargnent aux patients beaucoup d'effets secondaires ou de complications. Les médicaments Les médicaments anticoagulants oraux directs, par exemple, sont considérés comme des produits coûteux, mais ont un niveau d'efficience élevé là où d'anciens traitements anticoagulants, certes moins coûteux, entraînaient environ 5 000 décès chaque année. le coût d'un médicament ne peut être considéré comme un indicateur pertinent pour déterminer sa prise en charge, ou non, par l'assurance maladie, ne serait-ce qu'en raison de son caractère incomplet le coût des accidents, des hospitalisations, des soins de suite ou de la prise en charge d'un handicap provoqué par la prise d'un traitement, n'est pas comptabilisé dans le prix unitaire d'un médicament à l'achat en officine. La seule efficience d'un produit ou d'une prestation ne peut pas, et ne doit pas, être considérée comme une variable d'ajustement. La santé est un service public. Les besoins de santé ne doivent pas être subordonnés à des logiques de financement. Au contraire, c'est le financement qui doit être adapté aux besoins de santé. vous propose d'adopter cet amendement, qui vise à répondre à l'objectif d'une plus grande efficience des prescriptions, tout en assurant une meilleure sécurité juridique et une meilleure prise en compte de la valeur ajoutée médicale.

publique. La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit dans la partie législative du code de la santé publique l'obligation, pour le médecin, d'inscrire sur l'ordonnance la mention « non substituable non substituable » sous forme exclusivement manuscrite. À l'heure où les médecins sont fortement incités à informatiser les cabinets médicaux et où des expérimentations ont lieu sur les prescriptions électroniques, il n'est pas concevable d'obliger les médecins, pour chaque ligne de prescription, à porter la mention « non substituable substituable » sur l'ordonnance de façon manuscrite.

-et fixe également sa composition. Le second article arrête la procédure des tarifs et la classification des équipements matériels lourds. Il précise que le directeur général de l'UNCAM peut établir unilatéralement les tarifs et la classification des équipements lourds. Ces deux articles sont très préjudiciables à l'activité radiologique, privée ou publique, en ce qu'ils rompent avec les principes de la négociation conventionnelle.

On va aboutir à une diminution de l'utilisation des appareils les plus sophistiqués. Quand on interroge le SNITEM, le syndicat

Même s'il s'agit d'une procédure de dernier recours, et donc exceptionnelle, par cohérence avec sa position passée, la commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement. loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 que vous souhaitez supprimer créent les conditions d'une révision régulière des forfaits techniques des équipements lourds d'imagerie médicale. Il s'agit de mieux prendre en compte les innovations techniques et organisationnelles dans la fixation des tarifs. nous semble très judicieux, et je souhaite que la commission réunissant l'ensemble des acteurs concernés soit mise en place. Dans le cadre de cette procédure, le pouvoir des partenaires conventionnels pour fixer les différentes composantes des tarifs des forfaits techniques

L'objectif de ce dispositif est triple : lutter contre le gaspillage, car « chaque Français conserve en moyenne 1,5 kilogramme de médicaments non utilisés dans son armoire à pharmacie », limiter l'automédication et réduire le déficit de la sécurité sociale. Dans un contexte de crise économique, et au regard de la nécessité urgente de trouver de nouvelles ressources pour la sécurité sociale comme de faire des économies durables, il nous a paru nécessaire d'accélérer la mise en oeuvre du dispositif adopté voilà un an et de le généraliser.

Déjà en place en Angleterre ou en Allemagne, la délivrance de médicaments à l'unité peine à se développer en France. Pourtant, trois candidats à l'élection présidentielle de 2017, dont M. Emmanuel Macron, ont préconisé, dans leurs programmes, la vente des médicaments à l'unité. En campagne à Nevers, en janvier 2017, l'actuel Président de la République a affirmé que le passage au médicament à l'unité est un « impératif sanitaire, une nécessité économique et une évidence environnementale ». Il ajoutait : « Une expérimentation a déjà été lancée. Mais il faut aller beaucoup plus vite. Cela demandera une adaptation importante pour les industriels et les pharmaciens. » Si certains préfèrent faire des économies en déremboursant, il est préférable de faire des économies en déployant de nouvelles manières de dispenser les médicaments », avait également indiqué le candidat sur Twitter. Madame la ministre, à quelle vitesse nous mettons-nous « en marche » dans ce domaine ?

voire de pharmacovigilance. Pour les pharmaciens, la préparation des doses à administrer pour certains publics, notamment les personnes âgées, serait une évolution plus intéressante.

Les expérimentations ont eu lieu. Nous venons de recevoir le rapport final ; nous allons voir comment utiliser ces résultats.

sans surprise, en tout cas ! -, que le dossier n'a pas été préparé par le ministère précédent. Mme la ministre ne peut pas nous apporter de réponse aujourd'hui, elle n'était pas aux affaires voilà un an ...

praticien hospitalier d'être détaché dans un établissement de santé privé non lucratif, avant l'accomplissement de la période de service de trois années exigée par le code de la santé publique, a été supprimée par le décret du 29 septembre 2010. Désormais, aucun praticien ne pourra être détaché dans un établissement de santé privé non lucratif avant la réalisation de trois années de service. Ces restrictions ont profondément fragilisé l'offre de soins assurée par les établissements privés à but non lucratif, avec le concours des praticiens hospitaliers détachés. proposons donc d'insérer un nouvel article dans le code de la santé publique permettant aux praticiens hospitaliers d'être détachés à l'issue de la fin de la période probatoire d'un an d'exercice effectif.

la grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice libéral. Une telle situation, aggravée par un faible, met en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, elle est même particulièrement alarmante et engendre des effets cumulatifs. En effet, le surcroît de travail lié au manque de personnel de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés. Ainsi

lequel prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation. Les modalités d'accomplissement de cette durée minimale seraient définies par les conventions nationales conclues entre les professionnels et l'assurance maladie.

vous avez entendu le mécontentement des dentistes et, dans une volonté d'apaisement, vous avez convoqué une nouvelle négociation conventionnelle, en repoussant d'un an l'entrée en vigueur du règlement arbitral concernant l'application des plafonnements, la revalorisation tarifaire, la réévaluation des actes et, par voie de conséquence, le déclenchement de la clause de sauvegarde. Que veulent les dentistes ? Ils vous l'ont dit, ils ne veulent pas que le règlement arbitral vienne de nouveau menacer l'équilibre économique de leur profession et, ainsi, réduire leur capacité à fournir des soins de qualité à la population. Ils ne veulent pas que le règlement arbitral s'arrête à la seule revalorisation des consultations, en contrepartie du plafonnement du prix des prestations et à la mise en place d'une clause de sauvegarde. Ils veulent en finir avec les ajustements de circonstance. de circonstance. Ils veulent qu'une véritable discussion s'engage pour refondre un modèle qui n'a pas évolué depuis trente ans. Et ils veulent surtout qu'il soit tenu compte, dans le système de régulation et d'encadrement, des techniques innovantes et des enjeux de la prévention. Dans ce dossier, où les relations devaient être rénovées, nous pouvons saluer votre esprit de dialogue. D'ailleurs, vous avez écouté les dentistes, en donnant déjà, en vue de la négociation, des orientations très précises concernant la prévention bucco-dentaire. Nous nous interrogeons toutefois sur le résultat des négociations, dans la mesure où ces dernières sont rouvertes dans un cadre de réflexion obsolète, au regard des progrès de la science et des besoins de santé des Français, et, surtout, toujours sous la contrainte d'un éventuel nouveau règlement arbitral. Les négociations sont en cours. La voie conventionnelle doit être privilégiée, vous l'avez dit. C'est pourquoi la procédure du règlement arbitral,

La procédure arbitrale est en effet prévue pour être applicable, en cas de blocage des négociations, à l'élaboration d'une nouvelle convention et non à la mise en oeuvre d'un avenant ponctuel. aujourd'hui dans une situation différente, après la fronde des chirurgiens-dentistes face à ce qu'avait mis en place le gouvernement précédent. Madame la ministre, vous vous êtes engagée à relancer les négociations et le dialogue avec les professions de santé. Pour autant, je crains qu'il ne soit trop tard pour supprimer purement et simplement ce règlement arbitral, dans la mesure où certaines de ses mesures, notamment celles qui sont relatives à la prise en charge des soins pour les personnes fragiles, sont déjà entrées en application. il n'a pas semblé pertinent à la commission de mettre en place un moratoire s'agissant des relations entre l'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, alors même que tout devrait être fait pour restaurer la confiance et le dialogue dans les voies de droit commun. Les professions de santé dentaire sont

En second lieu, la rédaction proposée ne comprend pas de mécanisme de désignation en cas de désaccord entre l'assurance maladie et les organisations syndicales. sécurité sociale précise que, en cas d'opposition, l'arbitre est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Si je comprends le souhait de ne pas contourner les professionnels, il me semble cependant qu'il faut également pouvoir sortir d'une situation de blocage.

sur l'article. Madame la ministre, vous avez indiqué que le tiers payant ne pourrait pas être généralisé à l'ensemble de la population dans le calendrier et les conditions fixés en raison de problèmes techniques.

des affaires sociales, sur lequel vous vous appuyez, est beaucoup plus nuancé que ce que vous avez dit. On ne peut pas tirer si rapidement un trait sur un tel progrès social. Rappelons que le tiers payant s'adresse non pas aux personnes les plus démunies, mais essentiellement aux classes intermédiaires, dont les salaires sont un peu plus élevés.

et pour 64,5 % des femmes enceintes, selon la direction générale de la santé. On est donc très attentif au déploiement de cet outil, mais dans une logique d'appropriation par les médecins, conformément à la volonté de ne pas aggraver leur charge administrative. En tant que patient potentiel, je préfère que le médecin s'occupe de moi pour ce

Corinne Féret. Madame la ministre, je l'ai dit au cours de la discussion générale, vous avez tort d'abandonner le caractère obligatoire de la mise en place du tiers payant.

L'IGAS a confirmé que la mise en place du tiers payant obligatoire au 30 novembre 2017 était « irréaliste ». Pour notre part, nous avons toujours souligné la complexité, pour les médecins, d'appliquer ce tiers payant, eu égard au nombre d'organismes complémentaires.

les patients qui ne peuvent pas accéder au tiers payant généralisé sont ceux qui ont une complémentaire santé, en raison de la difficulté technique d'accéder à 250 complémentaires différentes, avec des niveaux de contrats très hétérogènes.

M. Yves Daudigny, pour explication de vote. Madame la ministre, nous ne sommes pas en désaccord sur tout. Je l'ai indiqué, nous ne réfutons pas tous les arguments que vous avez avancés. Là où nous ne sommes pas en phase, c'est sur la définition de l'objectif. Vous écrivez, à l'article 44 : « Cette concertation doit permettre de fixer le calendrier selon lequel le tiers payant intégral pourra être généralisable à tous les assurés. L'accord se serait fait si vous aviez mentionné « selon lequel le tiers payant intégral pourra être généralisé à tous les assurés ». Vous auriez même

la dispense intégrale de paiement. Il faut viser un système simple, à flux unique. Alors, madame la ministre, il n'y aura pas de perte de temps médical. Au contraire, il y aura gain de temps médical

Notre ancien collègue Jean-Pierre Bosino fut à l'initiative de cette proposition visant à réviser la liste des pathologies ouvrant droit au congé de longue durée pour les fonctionnaires. Pour rappel, le congé de longue durée est accordé aux agents de la fonction publique pour cinq pathologies : la tuberculose, la poliomyélite, les affections cancéreuses, les maladies mentales et le déficit immunitaire grave et acquis ou SIDA. Notre amendement tend à demander

pour mieux répondre aux besoins de la population. Vous le savez, en plus de trente ans, de nouvelles pathologies sont apparues, d'autres ont disparu, ce qui est tout à fait positif ; il faudrait donc en tirer les conséquences. Mme Touraine, ministre de la santé du gouvernement précédent, nous avait demandé d'attendre les conclusions des travaux des organisations syndicales sur la santé et la sécurité au travail. Ces travaux devaient

Le chantier de réforme des instances médicales de la fonction publique est engagé ; il est inscrit à l'agenda social 2017-2018 fixé par le ministre chargé de la fonction publique, Gérald Darmanin. Ce chantier nous donnera l'opportunité de remettre à plat les règles de gestion des divers congés de maladie des agents publics, pour la sclérose en plaques comme pour d'autres pathologies- vous avez raison, madame la sénatrice : certaines sont aujourd'hui mieux traitées que d'autres. plat permettra de faire évoluer cette liste et ces congés en cohérence avec les avancées thérapeutiques. C'est d'ailleurs ce que vous suggérez, madame Cohen. Pour cette raison, et parce que votre amendement me semble être un cavalier législatif, qui n'a pas vraiment sa place

de nombreuses études ont démontré que le dispositif de l'aide médicale de l'État n'était pas suffisamment efficient pour garantir un bon accès aux soins, que les ruptures étaient multiples dans les parcours de soins.

aux personnes en situation irrégulière, impliquerait de revoir l'un des principes sur lesquels est bâti le droit de la sécurité sociale. Cela conférerait à cette dernière une universalité inédite, par l'attribution du statut d'assuré social aux étrangers en situation irrégulière, alors même que la régularité du séjour constitue le discriminant entre assuré social et bénéficiaire de l'AME. En revanche, il est vrai qu'il faut peut-être améliorer en profondeur le pilotage des relations financières

Gouvernement ? Cet amendement à deux objets bien distincts : la couverture maladie des plus précaires et l'intégration de l'AME dans l'assurance maladie. Vous le savez, l'accès effectif aux droits des personnes les plus précaires

relèvent de deux logiques différentes. Je suis extrêmement attachée à l'AME, qui a pour objet de soigner des personnes démunies en situation irrégulière vivant sur le territoire. Elle relève, à ce titre, de l'action sociale et humanitaire financée par l'État. De plus, le panier de soins remboursés par l'AME diffère un peu du panier de soins de la sécurité sociale. Il ne donne pas accès, par exemple, aux cures thermales, ce qui paraît cohérent ! C'est normal ! Notre système de sécurité sociale, lui, est fondé sur les contributions obligatoires des assurés en contrepartie d'une couverture universelle face aux aléas de santé. Le rapport

Madame la ministre, je souhaiterais vous alerter sur les conditions de mise en oeuvre de la réforme des transports inter-établissements, qui cristallise le mécontentement de l'ensemble des acteurs hospitaliers ; nous les avons reçus. Vous le savez, cette mesure, prévue par la dernière loi de financement de la sécurité sociale, consiste à transférer la charge de cette dépense de l'assurance maladie aux établissements de santé, dans l'objet affiché de diminuer ce poste budgétaire par une responsabilisation des hôpitaux. Il semble cependant que le chiffrage proposé par la CNAM pour la détermination de l'enveloppe financière correspondante ne fasse pas- c'est là un euphémisme ! -consensus : les acteurs hospitaliers la jugent très significativement insuffisante. insuffisante. Ils ont souligné le risque d'incitation au contournement des règles qui pourrait résulter de l'application de cette réforme insuffisamment concertée. Les hôpitaux pourraient en effet être encouragés, en cas de besoin de soins relevant d'un autre établissement, à recourir à des sorties plutôt qu'à des transferts, afin de continuer à faire prendre en charge les transports correspondants par l'assurance maladie. Sans porter de jugement sur le fond de ces arguments, notre commission a estimé que les conditions n'étaient manifestement pas réunies pour l'application sereine de cette réforme. De nombreux amendements avaient d'ailleurs été déposés sur ce sujet, ce qui témoigne d'une inquiétude forte et partagée. J'aurais moi-même souhaité reporter cette réforme au 1 octobre 2019, afin de permettre un approfondissement de la concertation. Malheureusement, les règles de recevabilité financière des amendements ne l'ont pas permis. Madame la ministre, il m'a semblé important de il m'a semblé important de relayer ces inquiétudes. Vous pourrez peut-être les apaiser en apportant des précisions sur les orientations que vous fixerez pour la détermination de l'enveloppe budgétaire qui sera transférée au budget des établissements de santé pour la prise en charge des transports inter-établissements.

Les efforts d'efficience de ceux-ci sont ainsi absorbés par le dynamisme des dépenses de soins de ville. L'ONDAM exécuté se révèle éloigné de celui qui était initialement soumis à l'approbation du Parlement. Comme l'a constaté la Cour des comptes dans un récent rapport, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l'adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, mécanisme actuellement inexistant, à l'exception, nous le savons bien, des dépenses de médicaments. La Cour a ainsi réitéré sa recommandation d'instauration de dispositifs plus complets de suivi et de régulation infra-annuelle des dépenses de soins de ville.

la commission ? La commission est sceptique quant à l'opposition qui est souvent faite entre les soins de ville et les soins hospitaliers. Ce n'est qu'en créant les conditions d'une plus forte coopération et d'une meilleure complémentarité entre ces deux pôles

Je souligne d'ailleurs que les rapports d'activité de ce fonds ne sont plus disponibles en ligne ; ce n'est pas de nature à nous éclairer. Les professionnels que nous avons rencontrés lors des auditions ont mis l'accent sur l'investissement

Ils sont souvent accompagnés pour cela par l'Agence française de développement et la Banque publique d'investissement. La mise en place d'un établissement dédié à l'investissement immobilier des hôpitaux ne nous paraît pas nécessaire. Cependant, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

dans le cadre du modèle de la transition de la réforme du financement SSR sur le volet « Dotation modulée à l'activité ». L'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit la possibilité de mettre en place deux grilles tarifaires nationales, distinctes entre catégories d'établissements, concrétisées concrétisées par un premier arrêté ministériel en mai 2017. Ces tarifs nationaux « tout compris » correspondent à un périmètre de remboursement identique pour toutes les catégories d'établissements. Dès lors, et au regard de l'objectif de simplification du dispositif prévu à l'article 48 du projet de loi 2018, cet amendement a pour objet de fixer une échelle tarifaire unique pour l'ensemble des établissements SSR.

L'article 48 prolonge de deux ans le dispositif transitoire prévu en 2017 pour assurer une mise en oeuvre progressive des nouvelles modalités de financement des activités de soins de suite et de réadaptation. Ces réadaptation. Ces activités sont très hétérogènes, et les tarifs sont censés refléter des différences de coûts de prise en charge. Tout en partageant les objectifs de la réforme du financement des SSR, la commission avait regretté l'absence d'évaluation de ses effets sur les établissements.

Madame la ministre,

aux dépenses de personnel, aux frais d'approche- transports et taxes -, aux évacuations sanitaires, mais également à la mise aux normes des bâtiments en matière sismique et cyclonique. Les coefficients géographiques appliqués dans les outre-mer par la sécurité sociale aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l'Hexagone- 26 % pour la Guadeloupe et la Martinique ; 31 pour la Réunion et la Guyane -, ne compensent pas les charges pesant sur les hôpitaux. C'est ainsi que, chaque fin d'année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée aux établissements de santé. C'est la raison pour laquelle, en vue d'assurer un financement réaliste et adapté à la situation des outre-mer, cet amendement vise à préciser les critères sur lesquels reposent les coefficients géographiques.

Je souhaite un retrait de cet amendement, monsieur le sénateur. En effet, les surcoûts liés à l'insularité et l'éloignement géographiques sont d'ores et déjà intégrés dans le calcul du coefficient géographique. Cela inclut l'ensemble des éléments qui sont mis en avant, c'est-à-dire les surcoûts liés aux dépenses de personnel,

En réalité, on fait peser sur les malades une charge qui allège les dépenses de la sécurité sociale. Or, je le rappelle, même pour ceux qui ont des complémentaires, les cotisations à l'assurance maladie sont liées aux ressources, alors que les complémentaires ne le sont pas.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Je tiens à le rappeler, le forfait hospitalier, qui correspond à la participation des patients aux frais d'hébergement lors de leur séjour à l'hôpital, n'a pas été revalorisé depuis 2010. Cette augmentation de deux euros correspond donc à l'inflation cumulée de 2010 à 2017, en incluant 2018 par anticipation. Je précise également que la grande majorité des assurés sociaux n'auront pas à payer ce forfait journalier. D'une part, pour certaines catégories de patients, le forfait hospitalier est totalement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Je pense aux femmes enceintes,

la hausse totalement prise en charge par leur mutuelle. Il reste 5 % des Français qui n'adhèrent pas à une mutuelle. Mais tous les contrats de mutuelles couvrent le forfait journalier de manière illimitée. Il n'y aura donc pas de répercussion directe

tarifs. Je pense que la méthode choisie n'est pas la bonne. Le forfait hospitalier pèse déjà trop lourd pour un certain nombre de nos concitoyens hospitalisés.

s'inscrit dans le droit fil de l'intervention de Mme la ministre s'agissant des services de suite et de réadaptation.

une part des tarifs entre dans le budget des services de soins de suite et de réadaptation. Or il existe des différences considérables entre ces établissements selon les activités qu'ils pratiquent et, surtout, selon les méthodes qu'ils utilisent.

des services de suite spécialisés, ceux qui, notamment, traitent de l'obésité ou prennent en charge des réadaptations lourdes, pour des personnes qui sont complètement cassées et qu'il faut remettre sur pied le mieux possible. Tout cela n'est pas pris en compte, ce qui engendre des difficultés.

un point d'étape sur l'avancement de la réforme du financement des SSR est réalisé chaque année. L'année prochaine, un bilan de la première année de mise en oeuvre de cette réforme pourra être effectué et concernera l'ensemble des catégories d'établissements, y compris les soins de suite spécialisés. Pour ces raisons, votre amendement

Cet amendement vise à rendre publiques les décisions des agences régionales de santé, les ARS, en matière d'attribution des fonds aux établissements de santé. Il s'agit donc d'accroître la transparence du financement de l'assurance maladie et de permettre un accès libre aux données d'attribution des fonds publics.

Parlement, prévu dans un article du code de la santé publique. De surcroît, la mesure proposée ne fournirait qu'une information partielle dans la mesure où elle ne couvre pas l'intégralité des mesures relatives à la gestion du FIR.

Nous débattons depuis plusieurs jours de la santé des Françaises et des Français, ainsi que de l'accès aux soins en maintenant et en développant une qualité et une offre de soins partout sur notre territoire.

ne présentant, bien évidemment, aucun risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des personnels et des usagers est plus que jamais d'actualité. Si nous demandons un moratoire, c'est que le constat est plus qu'alarmant entre 1995 et 2005, près de 1 200 recompositions hospitalières ont eu lieu en France ; entre 1992 et 2003, 83 000 lits d'hospitalisation complète ont été supprimés, soit 15 % des capacités installées ; 380 établissements- 11 % des établissements existants en 1992 -ont été supprimés ou regroupés ; le nombre de lits a baissé dans le secteur public de façon beaucoup plus importante que dans le secteur privé, en pourcentage comme en volume. Le nombre de maternités a, quant à lui, chuté de 60 % en trente sans parler des conséquences que cela a entraîné sur les centres d'interruption volontaire de grossesse : en dix ans, ce sont 130 centres qui ont été fermés. Dans mon département, une maternité de secteur 1, celle d'Ivry-sur-Seine, a été fermée au profit de celle de secteur 2 du Kremlin-Bicêtre.

il est absolument indigne de laisser ouverts des hôpitaux de proximité qui n'ont pas les bons plateaux techniques, qui ne disposent pas de praticiens formés et où aucun d'entre nous n'irait se faire soigner

Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens s'inscrivent trop souvent dans une logique comptable. Surtout, cet article franchit un cran supplémentaire, en permettant à ces contrats de déroger aux conventions collectives des salariés des EHPAD. La suppression de l'opposabilité des conventions collectives de travail nous semble tout à fait incompréhensible. Je le sais, le Gouvernement justifie ce choix au motif que les conventions collectives collectives entreraient en contradiction avec les CPOM, surtout avec leur logique de financement. Alors que le secteur est déjà marqué par une grande précarité, cette mesure nous paraît injuste pour les personnels qui subissent des conditions de travail très difficiles et non reconnues ; je reviendrai sur ce point Enfin, cette mesure contribuera au démantèlement du statut collectif des personnels du secteur social et médico-social.

je ne peux être que défavorable à cet amendement, qui vise à mettre un terme aux réformes engagées dans le secteur médico-social. Je rejoins totalement mes collègues du groupe CRCE sur le constat quant aux carences du secteur, mais pas du tout sur le diagnostic.

seulement partielle de places. Cet amendement tend à sécuriser le dispositif pour les places effectivement ouvertes par les établissements qui ne pourront se voir menacer de caducité.

les autorités. Alors que, aujourd'hui, l'autorisation ne peut être retirée qu'en totalité, il sera demain possible de ne la retirer que partiellement si une partie de l'établissement est ouverte dans les délais.

de moyens de type EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec le conseil départemental et l'agence régionale de santé, l'ARS, et à l'obligation de se conformer au dispositif de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses,

Concept créé par la Mutualité sociale agricole, les MARPA, établissements relevant de la réglementation médico-sociale, constituent une solution d'hébergement intermédiaire entre le domicile et l'EHPAD. Outre l'intérêt que représente cette offre pour les seniors du milieu rural et périurbain, ces structures bénéficient à plus d'un titre aux territoires sur lesquels elles sont implantées. les MARPA forment un réseau de près de 200 maisons en fort développement en métropole, mais également hors métropole. Chaque projet de maison reçoit le soutien financier d'une caisse de la Mutualité sociale agricole et résulte de partenariats avec les collectivités territoriales. Les MARPA, qu'elles soient sous le statut de résidence autonomie, ne perçoivent pas de crédits d'assurance maladie. En outre, le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se fait comme à domicile. Il semble donc injustifié que le CPOM tripartite et l'EPRD s'imposent

Cette possibilité de dérogation, qui s'adresse essentiellement aux petites unités de vie non médicalisées, leur permet d'échapper au droit commun de la tarification et de la contractualisation pluriannuelle. les petites unités de vie médicalisées, qui ont une identité de gestionnaire avec des EHPAD, il me paraît plus sain pour le maillage et la viabilité de ces structures de maintenir l'obligation de CPOM et d'EPRD. Je souhaite néanmoins demander l'avis du Gouvernement, notamment sur la question des petites unités de vie déconnectées des EHPAD en zones rurales ou isolées.

Les établissements et services chargés de la prise en charge du handicap auraient l'obligation de contracter un CPOM unique à la triple condition d'une identité de gestionnaire, de ressort territorial et de mode de tarification.

médico-social. Ensuite, il convient de laisser une marge de manoeuvre aux ARS et aux conseils départementaux pour qu'ils jugent de l'opportunité et du bien-fondé de ces regroupements, au regard notamment des situations particulières. Enfin, compte tenu des réformes lancées à partir de 2016 sur le secteur des EHPAD et du handicap,

Ensuite, si nous voulons que le secteur médico-social entame sa mue nécessaire, il nous faut absolument responsabiliser les gestionnaires d'établissements et leur donner des marges de manoeuvre. L'avis est donc défavorable.

Le pôle d'activités et de soins adaptés, le PASA, est un espace d'accueil pour les résidents en EHPAD souffrant de troubles cognitifs consécutifs notamment à une maladie neurodégénérative, parfois associée à un syndrome démentiel, afin de conserver les acquis.

qui ouvre le forfait global de soins et les financements complémentaires aux établissements d'accueil de jour. Par ailleurs, il formule une possibilité déjà ouverte aux gestionnaires des EHPAD assurant des accueils permanents, qui reçoivent des financements complémentaires au titre des PASA. La commission demande le retrait

des organismes gestionnaires. La mesure de suppression de l'opposabilité des conventions collectives de travail aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, annoncée sans qu'une concertation avec les acteurs du secteur ait eu lieu, risque de fragiliser l'exercice des missions des associations au service des personnes accueillies et accompagnées. Bien que cette suppression de l'opposabilité soit compensée par la garantie de la libre affectation des excédents d'exploitation éventuels, il est essentiel que les pouvoirs publics n'affaiblissent pas le secteur du médico-social, qui accompagne au quotidien

commission ? Le dispositif de cet amendement, que je rejoins dans son principe, a l'inconvénient d'être un peu prématuré. Je le rappelle, le dispositif de l'appartement de coordination thérapeutique se présente comme un dispositif médico-social de suivi rapproché de personnes en situation de très grande vulnérabilité physique ou psychologique. Comme il fonctionne sur le modèle du gestionnaire de cas, son extension en service d'intervention à domicile, qui suppose une forme de généralisation, ainsi qu'une modification

les réponses apportées ne me satisfont pas. Il s'agit d'une urgence : dès la fin de cet hiver, il y aura de nouvelles expulsions de personnes atteintes de pathologies lourdes et en situation extrêmement précaires. Ce n'est plus une affaire comptable, c'est une affaire d'humanité.

Ces données arrivent dans un contexte particulièrement tendu : convergence à la baisse des budgets de nombreux établissements ; arrêt des contrats aidés ; rapport parlementaire

une « mission flash » sur la situation des EHPAD, qui a confirmé ce constat négatif. C'est dans ce contexte que la réforme de la tarification se met en place et provoque des inquiétudes légitimes, notamment dans les EHPAD publics. Les personnes âgées les plus dépendantes sont d'ailleurs affectées du

la perte subie notamment par les EHPAD publics au titre de la dotation dépendance serait en quelque sorte compensée par l'augmentation du forfait soins et les mesures en faveur du financement d'une infirmière de nuit. Mais les EHPAD publics les ont déjà mis en place ! Au final, le rapporteur de la commission des affaires sociales nous a indiqué- il l'a confirmé lors de l'examen de ces dispositions par la commission

défavorable à l'idée de moratoire ! La réforme de la tarification des EHPAD vise à modifier le système de la reconduction historique, qui ne satisfait pas aux objectifs de la prise en charge adaptée et de la bonne gestion des deniers publics. que, au vu des augmentations tarifaires que connaissent globalement les EHPAD- j'insiste, madame la ministre, sur le terme « globalement » -depuis la réforme des forfaits soins et autonomie, c'est à un manque à gagner criant que le dispositif les condamnerait.

J'ai néanmoins été alertée tout l'été par différents élus sur les risques encourus par certains EHPAD. Aussi, nous avons donc mis en place au sein du ministère un comité de suivi, qui s'est réuni pour la première fois le 25 septembre dernier. Ce comité fait un état des lieux régulier des difficultés rencontrées, qui remontent du terrain. est de la philosophie de la réforme, il faut continuer en ce sens. C'est une bonne réforme, qui distingue les soins, la dépendance et l'hébergement. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. Vous le savez, 397,9 millions d'euros de financements supplémentaires seront alloués aux EHPAD sur la période de sept ans.

Bien que les prévisions pour le tarif dépendance laissent apparaître un solde négatif de 65,6 millions d'euros pour l'ensemble des 3 400 établissements publics sur sept ans,

de 100,2 millions d'euros de financements supplémentaires à l'issue de la période de convergence. Selon nos chiffres, seuls 2,9 % des EHPAD, tous secteurs confondus, cumulent les effets d'une convergence négative sur leur forfait soins et dépendance. Pour ces établissements, nous dégageons une enveloppe de 28 millions d'euros, qui pourra être utilisée spécifiquement pour accompagner ces établissements.

ce secteur, qui devra rédiger une charte nationale d'engagement pour la qualité de vie au travail pour les employeurs publics et privés des EHPAD. Un guide à destination des EHPAD sur la qualité de vie au travail, piloté par l'Agence va être réalisé. Des instructions aux ARS seront données pour intégrer la dimension de la qualité de vie au travail au sein des CPOM. Tout un tas de mesures d'accompagnement se mettent en oeuvre, pour tenir compte des remontées du terrain. En conséquence, l'avis est défavorable.

au problème regrettable de la sous-consommation des crédits relatifs à l'APA 2. Regrettable, ce problème l'est à deux égards : pour les départements, qui sont dans la situation paradoxale de ne pouvoir dépenser des crédits dont ils ont grandement besoin besoin ; pour les réserves de la CNSA, qui se trouvent artificiellement gonflées par ces recettes inemployées. En proposant de fusionner le reliquat non consommé de l'APA 2 et le montant de l'APA 1, c'est une mesure de clarification financière et de soutien aux départements que la commission

MAIA. Cette mesure, qui rejoint les préconisations du Conseil économique, social et environnemental, mais aussi certaines pratiques de terrain déjà constatées, dont les retombées semblent très positives, a pour objet d'encourager le rapprochement des structures d'accompagnement des personnes âgées, dans un double objectif de mutualisation des coûts et de lisibilité des services pour les publics concernés.

Dans mon département, on a choisi de compenser le désengagement des emplois de l'État, non pas par une mise à disposition de fonctionnaires, mais par une augmentation de la dotation. Avec cet amendement, le choix serait fait de privilégier la mise à disposition de personnel

La mutualisation de la PCH dans le cadre de ces logements autonomes ou semi-autonomes est un pas nécessaire qu'il nous faut franchir, ne serait-ce qu'avec le souci d'assurer une sécurité juridique aux personnes qui la pratiquent déjà. Je salue l'initiative de notre collègue Philippe Mouiller. C'est pourquoi j'émets un avis favorable. du Gouvernement ? Monsieur le sénateur, cet amendement vise à introduire la possibilité d'une mutualisation de la PCH entre plusieurs personnes handicapées dans le but d'optimiser les aides et l'aménagement des logements. logements. Il manifeste le soutien au développement de l'habitat inclusif ; c'est un souci qui est partagé, notamment par Sophie Cluzel, qui l'a rappelé en conseil des ministres le 7 juin dernier et qui fait de ces actions une priorité du quinquennat. Les services de l'État sont d'ores et déjà engagés, en coopération avec le secteur associatif, dans une démarche nationale en faveur de l'habitat inclusif. Des premières mesures concrètes d'encouragement ont été mises en place, avec une aide spécifique forfaitaire d'un montant de 60 000 euros attribuée par les ARS. L'Observatoire de l'habitat inclusif, qui est le lieu de référence en matière d'habitat inclusif pour les personnes âgées et les personnes handicapées, a été installé le 10 mai dernier et produira, à l'occasion de la journée nationale de l'habitat inclusif le 30 novembre prochain, un guide d'aide au montage de projets. Pour la suite, si les travaux conduisent à identifier des obstacles juridiques au développement de ces formes d'habitat, nous veillerons à les lever, en utilisant au besoin les voies législative- ce que vous proposez -et réglementaire. À ce stade, suivant les recommandations du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de novembre 2016, le Gouvernement a élaboré une fiche relative à la mise en commun de la PCH qui en explicite d'ores et déjà les modalités de réalisation, afin de faciliter les projets d'habitat inclusif. L'objet de votre amendement est donc satisfait.

Laurence Cohen, sur l'article. L'article 51 prévoit la suppression de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, l'ANESM, et la reprise de ses compétences par la Haute Autorité de santé, La convention nationale des associations de protection de l'enfant s'est inquiétée des conséquences de cette fusion et de la prise en compte spécifique des aspects sociaux et médico-sociaux, qui pourraient sortir rapidement des préoccupations de la Haute Autorité de santé. La crainte est donc grande que la HAS, qui a une histoire et un champ de compétences déjà vaste, ne soit pas en mesure d'appréhender toutes les spécificités d'un secteur qui comprend des structures de protection de l'enfance, de lutte contre les exclusions, d'accueil des demandeurs d'asile, de personnes âgées ou en situation de handicap et des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Par ailleurs, l'absence de concertation avec les personnels semble susciter chez eux une forte inquiétude pour leur avenir, alors qu'ils ont appris la décision de fusionner la HAS de loi de financement de la sécurité sociale. Vous avez répondu à nos collègues députés que cette décision était prévue depuis de nombreuses années. Pourtant, la concertation en amont ne semble pas avoir eu lieu, ce qui est fortement regrettable. Bref, cette fusion ne nous convainc pas ; au contraire, elle nous inquiète.

Il est défendu. Quel est l'avis de la commission ? la fusion des deux agences. Il paraît légitime, en effet, que l'intégration de l'ANESM entraîne un ajustement de la composition du collège de la HAS. Néanmoins, le dispositif pose plusieurs problèmes d'ordre juridique. Tout d'abord, la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale a, aujourd'hui, une existence seulement réglementaire, et non législative, et sa mission est consultative. Il serait donc curieux d'ajouter ce comité à la liste des autorités constitutionnelles qui sont chargées de nommer les membres du collège de la HAS. ces autorités sont libres de leur choix de désignation, et rien ne les empêchera d'adapter la composition du collège en nommant, la prochaine fois que cela sera prévu, un représentant du secteur médico-social. Enfin, cet amendement prévoit que le membre supplémentaire du collège ne sera pas rémunéré. Or les membres actuels du collège perçoivent un traitement ou une indemnité en fonction de leur statut d'actif ou de retraité, et il n'est pas possible de prévoir un régime distinct pour le membre supplémentaire. Pour toutes ces raisons,

les constatations réglementaires effectuées par la commission, je voudrais rassurer le secteur médico-social à propos de la fusion entre la HAS et l'ANESM, qui est dans les tuyaux depuis de nombreuses années. En effet, lorsque j'avais pris la présidence de la HAS, il y a un an et demi,

pour tout le secteur social et médico-social ; je pense que cela sera évidemment fait. Dans ces commissions d'experts siégeront toutes les parties prenantes du secteur,

de leurs connaissances pour améliorer le champ de compétences des uns et des autres. Selon moi, il n'y a pas lieu d'inscrire quoi que ce soit dans la loi. Une nouvelle commission spécialisée sera créée

je souhaite vous parler de démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, depuis qu'elle a été consacrée par le Sénat, comme par l'Assemblée nationale, dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, repose essentiellement sur la reconnaissance de droits individuels et la représentation des usagers dans les instances de santé. Au-delà de ces éléments, c'est l'implication individuelle et collective des patients et des usagers dans les soins et la santé qui doit, à son tour, faire l'objet de nos préoccupations. nombreux pays la pratiquent, qui ont pris une avance notable dans la promotion d'attitudes nouvelles favorables à cette implication, sous la terminologie de participation ou de partenariat. C'est la partie que notre pays a un peu délaissée pour se concentrer sur les droits et procédures. Cependant, les changements d'attitudes dans le soin et la santé, tant des patients que des professionnels du soin, doivent découler non pas nécessairement de l'édiction de droits et de procédures, mais plutôt de recommandations et d'actions que la Haute Autorité de santé peut légitimement promouvoir, promouvoir, au titre de son indépendance et de sa légitimité scientifique. Il est proposé que les recommandations et les actions de la Haute Autorité de santé dans le domaine de la démocratie sanitaire puissent bénéficier des ressources du Fonds national

puisque le dernier alinéa du III de l'article L. 221-1-3 prévoit que « le fonds peut également participer au financement [ ...] d'organismes publics développant des activités de recherche

du Gouvernement ? Si la HAS intègre évidemment les acteurs de la démocratie sanitaire au sein de ses instances-

continuité des gouvernements précédents. Les victimes en seront malheureusement encore les personnels soignants et les assurés sociaux. C'est pourquoi nous voterons contre cet article.

elles atteint 800 millions d'euros. Au regard des grandes difficultés que rencontrent les établissements de santé, notamment l'hôpital public, nous souhaitons que cet écart soit comblé

Les dépenses de soins de ville devraient être dynamiques en 2018, avec une croissance tendancielle évaluée à 5,1 %. Le rapprochement des objectifs de dépenses entre ville et hôpital risquerait donc de conduire en exécution à un dépassement de l'ensemble de

Les ressources qui seront apportées aux établissements de santé permettront de financer l'investissement à hauteur de 400 millions d'euros, l'innovation, par la « liste en sus », à hauteur de 600 millions d'euros et des mesures nouvelles à hauteur de 200 millions d'euros.

soit une progression de 2,1 %, identique par rapport à 2017 si l'on ne tient pas compte de l'augmentation du forfait hospitalier. Je rappelle que, la semaine dernière, le Sénat a adopté le projet de loi de programmation des finances publiques prévoyant de réduire de 4 milliards d'euros le budget de la santé chaque année, avec un objectif national de dépenses pour l'assurance maladie dont la progression est maintenue à 2,3 % sur la période 2018-2022, tandis que les dépenses naturelles de la santé- nous l'avons dit et écrit ! -sont de l'ordre de 4,7 %. Cela signifie que le Gouvernement, suivant en cela les directives de la Commission européenne, a décidé de nous imposer une réduction des dépenses de la sécurité sociale pour 2018, mais aussi pour 2019 et, encore, pour 2020.

en espérant que les générations ultérieures trouveront les moyens de rembourser la dette. Il me paraît donc impératif- j'aurai toujours en ligne de mire ce que nous devons aux générations futures -de réduire la dette que nous laisserons à nos enfants.

réponse aux besoins liés au vieillissement de la population et aux polypathologies que nous observons actuellement. Il ne faut pas confondre l'augmentation des dépenses de santé avec l'augmentation des besoins.

Le scrutin est ouvert.

Elles sont actuellement subsidiairement et solidairement responsables en cas d'infraction de travail dissimulé : nous souhaitons qu'il en soit de même en cas de fraude aux cotisations sociales. Par cet amendement, nous proposons donc d'étendre ce principe au cas d'infraction de non-paiement des cotisations sociales. Il s'agit d'un outil de lutte contre la fraude patronale dont il serait dommage de se priver, tant cette fraude peut s'avérer coûteuse pour les deniers publics, dans une mesure d'ailleurs incomparablement plus importante que celle dont on discutera dans un instant. le rapport annuel de la Cour des comptes sur la sécurité sociale publié le 17 septembre 2014 indique que le montant des irrégularités et fraudes patronales, toutes branches confondues, a atteint, en 2012, un niveau record, entre 20,1

L'objectif est d'accentuer la lutte contre la fraude sociale. Cette lutte a déjà été largement renforcée au cours des dernières années. la fraude aux différentes prestations sociales- famille, vieillesse, assurance maladie -s'élève à 672 millions d'euros par an, soit 3 % de la fraude totale. Pour rappel, selon la Délégation nationale de lutte contre la fraude, la fraude fiscale représente, quant à elle, plus de 21 milliards d'euros Madame la ministre, vous avez parlé de gabegie : voilà une source où puiser ! Quant à la fraude patronale, elle s'élève chaque année à plus de 20 milliards d'euros. Il nous

à 4 milliards d'euros. Nous ne nions pas que certaines personnes malintentionnées perçoivent des prestations auxquelles elles n'ont pas droit, mais nous savons également -le rapport du défenseur des droits rendu public en septembre dernier dénonce ce fait -que cette chasse entraîne de véritables dérives, des stigmatisations et a des conséquences désastreuses pour certaines personnes de bonne foi. Nous reviendrons sur ce point lors de la présentation de notre prochain amendement. Madame la ministre, vous avez insisté, à l'Assemblée nationale, sur le fait que cet article permettait également de cibler les fraudes de certains professionnels de santé, vous défendant ainsi de stigmatisation. Certes, mais cela n'enlève en rien au fait que cet article, en l'absence d'un article relatif à la fraude patronale, par exemple, est particulièrement orienté politiquement et ne permettra pas, en outre, de remplir davantage les caisses.

En cas de méconnaissance involontaire des obligations déclaratives, la personne sera en effet invitée à rectifier son erreur après que l'organisme lui aura rappelé la règle applicable. Cette harmonisation, rappelée notamment par le défenseur des droits, permet ainsi de disposer d'un dispositif juridique

de relever la pénalité financière dont doivent s'acquitter les destinataires du droit de communication n'ayant pas satisfait aux demandes de l'organisme concernant des personnes non identifiées.

Le Gouvernement partage bien entendu votre souhait de lutter contre la fraude, mais cet amendement pose deux difficultés. D'une part, l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit déjà des plafonds de pénalités financières en cas de fraude. S'agissant de fraude commise en bande organisée, le plafond est de 300 % des sommes indûment remboursées, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale. L'adoption de votre amendement doublerait donc le plafond existant. part, le dispositif du droit de communication non nominatif créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 s'inspire du dispositif prévu en matière fiscale par l'article 1734 du code général des impôts. La sanction forfaitaire est du même montant- 5 000 euros -, dans un souci d'harmonisation avec le code général des impôts. Pour ces raisons, on peut considérer que votre amendement est déjà largement satisfait et que ses dispositions n'amélioreraient pas la cohérence et l'efficacité de la politique de lutte contre la fraude.

amendement a pour objet de permettre aux caisses de sécurité sociale du régime agricole de mettre en oeuvre, dans les mêmes conditions que les organismes de recouvrement du régime général, la procédure de saisie conservatoire prévue par le code de la sécurité sociale. est précisé que cette procédure peut s'appliquer non seulement lorsque les constats de travail dissimulé sont dressés par les URSSAF et les autres corps de contrôle, mais également dans le cas où ces constats sont réalisés par les agents de contrôle de la

Dans le prolongement du débat que nous venons d'avoir, nous reprenons ici l'une des propositions issues du rapport de Jacques Toubon, défenseur des droits, intitulé « Lutte contre la fraude aux prestations sociales : à quel prix pour les droits des usagers ? ». Ce rapport fait état de nombreux témoignages de bénéficiaires de prestations sociales qui, du fait d'un oubli, d'une erreur, se sont vus privés du jour au lendemain de leurs prestations. Les conséquences financières et sociales peuvent être évidemment très graves, notamment pour des personnes déjà précarisées. La rédaction du code de la sécurité sociale n'étant pas assez claire, il nous paraît essentiel qu'il soit écrit noir sur blanc que lorsque l'intention frauduleuse n'est pas avérée, aucune pénalité ne peut être infligée.

cet amendement ignore les apports de l'article 57, qui permet à une commission d'émettre un avis sur le cas contentieux avant que la pénalité ne soit prononcée. Cette instance devrait fournir des garanties suffisantes pour l'établissement de l'intention frauduleuse. Je souhaiterais néanmoins connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet. Quel est

: La parole est à M. Xavier Iacovelli. Cet amendement s'inspire du rapport parlementaire relatif à l'évaluation des politiques publiques en faveur de l'accès aux droits sociaux. Il vise à instaurer une mesure annuelle des taux de non-recours aux minima sociaux, aux minima sociaux, en imposant au Gouvernement la publication d'un rapport sur ce thème le 1janvier de chaque année. L'Observatoire des non-recours aux droits et services a dressé la typologie du phénomène du non-recours aux minima sociaux mais, aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de chiffrer ce taux de non-recours.

La persistance d'un taux élevé de non-recours à une prestation doit inciter les pouvoirs publics à réexaminer la façon même dont elle a été conçue et à s'interroger sur sa pertinence.

En outre, Mme Gisèle Biémouret et M. Jean-Louis Costes ont récemment présenté, au nom du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, un rapport très complet sur l'évaluation des politiques publiques en faveur de l'accès aux droits sociaux.

Je rappelle que, dans un rapport de 2013, la Cour des comptes estimait la fraude patronale aux cotisations sociales à 20 milliards d'euros. Parallèlement, la somme récupérée à la suite des interventions des agents de contrôle des URSSAF s'établit à 1,5 milliard d'euros, d'après le rapport d'activité pour 2016 de l'ACOSS. Sur cette somme, 555 millions d'euros sont recouvrés au titre du travail dissimulé. La présente demande de rapport vise à ce que nous puissions disposer d'une évaluation plus récente du montant de la fraude patronale aux cotisations sociales et de recommandations

En juin 2017, une évaluation objective et très précise a également été réalisée par les organismes sociaux sous l'égide du Conseil national de l'information statistique. À l'issue de ces travaux, sans doute les plus précis et les plus sérieux qui aient été conduits sur le sujet à ce jour, l'ACOSS a estimé que le montant de la fraude aux cotisations

Au cours de cette discussion, des dispositifs forts, essentiels, qui font quasiment consensus dans cet hémicycle, ont été votés. Je tiens à en évoquer deux. tout d'abord l'obligation vaccinale, nous ne le répéterons jamais assez : se protéger, c'est aussi être altruiste en protégeant les autres, en songeant au bien-être de tous et de toutes. La vaccination relève de la solidarité, d'une prise de conscience collective.

Toutes les familles ont leurs difficultés, c'est pourquoi je souhaite tout comme vous, madame la ministre, que soit lancée une grande réflexion sur la branche famille. Je regrette que le Sénat ne s'inscrive pas dans la même démarche. Pour cette raison, le groupe LREM votera contre la quatrième partie.